le secrétaire d'État, mes chers collègues, l'année 2020 qui s'achève et l'année 2021 qui vient sont très particulières du point de vue des relations, notamment financières, entre l'État et les collectivités territoriales. La crise sanitaire et économique a provoqué un effet ciseaux qui continuera de se faire sentir en 2021 et qui a justifié que le Parlement et le Gouvernement s'accordent sur des mesures de compensation, lesquelles doivent très certainement être approfondies. Je ne reviens pas davantage sur ces enjeux, que nous connaissons tous ici et dont Claude Raynal dira quelques mots. Je rappelle toutefois l'attachement de notre commission, madame la ministre, à ce que les collectivités locales soient en mesure d'être au rendez-vous de la relance. Cela implique un certain volontarisme de la part du Gouvernement- je sais que vous-même

et à 3,9 milliards d'euros en crédits de paiement, ce qui ne représente qu'une très faible part des transferts financiers de l'État aux collectivités territoriales, lesquels s'élèveraient à 104,4 milliards d'euros en 2021. La première caractéristique du budget qui nous est proposé est- une fois n'est pas coutume ! -sa stabilité. En effet, les hausses de crédits constatées tiennent, pour l'essentiel, à des mesures de périmètre.

La mission RCT porte une partie du plan de relance puisqu'elle permet de couvrir, à hauteur de 100 millions d'euros, les crédits de paiement afférents au milliard d'euros d'autorisations d'engagement consommées en 2020 au titre de la DSIL exceptionnelle votée dans le cadre de la troisième loi de finances rectificative. Cette dernière devait permettre de financer des projets relevant de trois priorités : la transition écologique, la résilience sanitaire et la rénovation du patrimoine. Au 15 octobre, 1 749 projets ont été programmés, pour un montant de 320 millions d'euros. Je le rappelle, sur l'initiative du Sénat, il avait été prévu que, à titre exceptionnel, ces crédits puissent financer des projets éligibles à la DETR. Ces derniers représentent à date environ 14 % des projets subventionnés.

de levier sur l'investissement local, qui doit être un pilier de la réponse à la crise économique. Mes chers collègues, comme les années précédentes, nous vous proposons d'adopter les crédits de la mission. le compte de concours financiers « Avances aux collectivités territoriales », qui voit notamment transiter le produit des impositions locales versées mensuellement par l'État aux collectivités territoriales : 111,5 milliards d'euros sont prévus à ce titre pour 2021. On constate une baisse de 1,3 % du montant de ces avances en 2021, cette baisse traduisant les effets de la crise sur les impôts locaux, après plusieurs années de dynamisme.

Le montant provisionné pour 2020 et 2021, de 2,7 milliards d'euros, pourrait être bien supérieur aux besoins. En effet, seuls quarante départements ont décidé de faire appel à ces avances à ce jour. Je rappelle que, sur que, sur l'initiative du Sénat, une clause de retour à meilleure fortune a été introduite : la période de remboursement ne démarrera qu'à compter de l'année suivant celle au cours de laquelle le montant des recettes fiscales de DMTO sera égal ou supérieur à celui qui a été constaté en 2019.

loi de finances pour 2020, notre commission des finances avait alerté sur ce que nous avions qualifié de « réforme cachée » dans la réforme de la taxe d'habitation, anticipant par là d'importantes variations des indicateurs de péréquation, compte tenu de la suppression de la taxe d'habitation. Sur ce point, les travaux du Comité des finances locales nous ont donné raison. Ce mécanisme de neutralisation, qui est une bonne nouvelle, fonctionne en deux étages. D'une part, il introduit une nouvelle méthode pérenne pour le calcul du potentiel fiscal afférent à la taxe foncière. D'autre part, il institue une fraction de correction du potentiel fiscal et des indicateurs financiers, laquelle permettra de neutraliser, par exemple, les effets du remplacement d'un produit potentiel par un produit réel. Cette fraction sera pérenne pour les départements et dégressive pour les autres collectivités. Le mécanisme proposé est donc à la fois une première solution et une invitation à engager une réforme ambitieuse de la péréquation.

Ce montant représentant plus du tiers des impôts locaux, nous assistons à une sorte de tsunami pour les finances locales, qui impose une incontournable et urgente réflexion dans trois directions

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, Charles Guené ayant dit l'essentiel, il me revient d'évoquer le reste L'année 2021 sera une année charnière pour les collectivités territoriales. À cet égard, j'aimerais à mon tour attirer votre attention sur quelques points de vigilance.

Trois régimes de compensation se distinguent. Le premier, le plus favorable, concerne Île-de-France Mobilités, qui bénéficie d'une compensation des pertes de versement mobilité calculée en référence à son taux de l'année 2019. Cette AOM percevra ainsi 1,2 milliard d'euros d'avances remboursables au titre de ses pertes de recettes tarifaires. Le deuxième régime s'applique aux AOM constituées en syndicat mixte, qui voient leurs pertes de versement mobilité compensées en tant que telles, en référence à une moyenne. Elles bénéficieront par ailleurs du versement d'avances pour tenir compte des pertes de recettes tarifaires. Enfin, le troisième régime s'applique aux EPCI qui exercent en propre la compétence d'AOM. Pour eux, la compensation est plus que sommaire

Malgré les apports du Sénat, je pense que le compte n'y est toujours pas. Se pose par ailleurs la question de la juste compensation des pertes de recettes fiscales subies par les collectivités territoriales. présent projet de loi de finances, le Sénat a adopté plusieurs mesures importantes afin de combler des lacunes du texte initial. Malgré la proposition de Jean-René Cazeneuve, le Gouvernement n'a pas reconduit en 2021 le mécanisme de garantie des ressources pour le bloc communal. Le Sénat s'en est donc chargé ! La question de la compensation des pertes de recettes tarifaires n'est toujours pas résolue à ce jour. J'ai conscience qu'elle pose certaines difficultés techniques puisqu'il faudrait pouvoir définir précisément le périmètre de la compensation en neutralisant les choix de gestion, très variables selon les communes. Ma conviction est néanmoins que nous devons collectivement trouver les moyens techniques, juridiques et politiques de les surmonter et engager un travail sur ce sujet dès que possible. Je dirai maintenant quelques mots dans la perspective de la discussion que nous allons engager aujourd'hui. Comme chaque année, le nombre élevé d'amendements qui a été déposé témoigne de notre souci commun d'agir en faveur des collectivités territoriales. Chers collègues, nous souhaitons attirer votre attention sur certains points. Je rappelle tout d'abord que le débat sur le niveau et le montant des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales a été tranché en première partie. Nous sommes donc désormais contraints de raisonner à enveloppe fermée : tout dispositif en faveur d'une catégorie de collectivités ne pourra être financé qu'au détriment des autres. Des choix politiques devront Par ailleurs, de nombreux amendements concernent le mode d'attribution des dotations de l'État, diverses propositions étant faites pour renforcer le rôle des commissions d'élus ou pour « départementaliser » la De façon constante, nous ne sommes pas favorables à de telles évolutions, qui alourdiraient les procédures sans toutefois apporter des solutions bien meilleures. Il s'agit là d'un débat que nous avons chaque année. Certaines années, nous parvenons à vous convaincre et les amendements en ce sens sont rejetés ; certaines années, nous n'y parvenons pas, et ces mêmes amendements sont adoptés. La seule chose qui ne varie pas, c'est leur absence totale dans le texte final ! Concernant plus spécifiquement la DETR, un article modifie les règles de calcul de l'enveloppe accordée aux départements, de rediriger la dotation vers les territoires les plus ruraux et de lisser l'évolution des montants d'une année sur l'autre. Il nous semble indispensable de revenir à l'objectif de la DETR, qui est de préserver et de soutenir l'investissement dans les territoires ruraux. Cette ambition, nous la partageons tous, me semble-t-il.

certaines simulations montrent que d'importantes variations des indicateurs et des dotations pourraient malgré tout se manifester, en dépit des dispositifs de neutralisation introduits à l'article 58. Nous avons toute l'année pour éventuellement corriger le mécanisme, ou à tout le moins nous convaincre de son intérêt. D'autre D'autre part, il me semble que les inquiétudes manifestées par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui ont été conduits à augmenter le taux de la taxe d'habitation entre 2017 et 2019 dans le cadre d'un pacte financier n'ont donné lieu qu'à de très rares réponses de la part de l'État. je rappelle que la réforme pourrait désinciter très fortement la construction de logements sociaux, ce qui serait désastreux. En effet, alors que, jusqu'ici, les communes et les EPCI percevaient une recette, même marginale, de taxe d'habitation, ils ne bénéficieront plus d'aucune recette à compter de 2021, alors même que les constructions neuves de logements sociaux sont exonérées de taxe foncière parfois pendant trente Il est absolument nécessaire d'agir. À cette fin, j'ai déposé un amendement en seconde partie du projet de loi de finances visant à transformer les actuelles exonérations de taxe foncière sur les constructions neuves de logements sociaux en dégrèvements. Certes, la mesure coûterait plus cher à l'État que ce que rapportait la taxe d'habitation acquittée par les ménages résidant dans des logements sociaux, mais le débat doit être posé : les communes et les EPCI perdent chaque année près de 525 millions d'euros de produit de taxe foncière au titre des logements sociaux et l'État entend les priver de plus de ressources encore, du fait de la suppression de la taxe d'habitation. De mon point de vue, ce n'est pas acceptable- ce n'est d'ailleurs pas accepté -, mais, pour l'instant, les propositions du Gouvernement tardent

les crédits inscrits au titre de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » connaissant une hausse significative pour 2021, la commission des lois n'a pu qu'émettre un avis favorable à leur adoption, sous réserve de l'adoption de trois amendements que je vous présenterai. S'il est S'il est effectivement heureux que, dans le contexte d'une crise sanitaire et économique inédite, l'État manifeste son appui à des collectivités territoriales dont les perspectives financières apparaissent plus incertaines que jamais,

Ces élans me semblent se manifester tout d'abord dans le contexte actuel des finances locales que nous connaissons tous, celui de la crise sanitaire, évidemment, au cours de laquelle le soutien financier de l'État aux collectivités a pu paraître faillible ou incomplet. Si ces critiques ne sont pas toutes dénuées de fondement, des manquements de l'État me semblent néanmoins totalement compréhensibles, en ce qu'ils peuvent être attribués à l'environnement de très grande incertitude financière dans lequel celui-ci agit. Il n'en va pas de même pour le second élément de contexte sur lequel je souhaite insister aujourd'hui : je veux parler du recul toujours plus prononcé du pouvoir fiscal des collectivités, qui voient les ressources sur lesquelles elles ont un pouvoir de taux ou d'assiette progressivement remplacées par des dotations ou des parts d'impôts nationaux. économiques proposée cette année ne fait pas exception à cette règle. Comment ne pas voir dans ce contrôle progressif des ressources des collectivités territoriales les prémices d'une recentralisation insidieuse, permettant à l'État de manier la subvention ou la dotation comme une « forme financière du contrôle », pour reprendre les mots du juriste Guy Braibant ? Ces élans recentralisateurs se manifestent également dans les modalités d'attribution par l'État des dotations de soutien à l'investissement. Je souhaiterais donc renouveler à cette tribune, au nom de la commission des lois, un appel à la plus grande vigilance sur l'association insuffisante et l'information parcellaire dont disposent les élus quant aux choix de l'État en la matière. Je vous sais, mes chers collègues, attentifs à cette question. J'en veux pour preuve la proposition de loi, déposée par notre collègue Hervé Maurey, pour laquelle notre collègue Bernard Delcros était rapporteur, et récemment adoptée par le Sénat, relative au renforcement des commissions DETR. Se fondant sur des constats que la commission des lois émet depuis plusieurs années, elle formule des solutions dont nous aurons de nouveau à débattre, et je m'en réjouis. Si elles sont perfectibles, les commissions DETR ont du moins le mérite d'exister

légèrement différente, tendant à mieux intégrer les élus locaux aux décisions de la DSIL. L'attribution d'une part significative de la DSIL au niveau départemental, selon des modalités proches de celles de l'attribution de la DETR, permettrait non seulement de mieux inclure les élus aux décisions de subvention, mais également de rapprocher celles-ci des besoins réels du terrain. À défaut, il pourrait être envisagé de créer une commission de suivi des investissements locaux.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, dans cette mission « Relations avec les collectivités territoriales » du projet de loi de finances (PLF) pour 2021, nous nous réjouissons que les concours financiers de l'État envers les collectivités territoriales soient en hausse de manière conjoncturelle, mais la baisse du montant des impôts économiques dont disposent les collectivités territoriales correspond structurellement à une perte d'autonomie grave. À court terme, avec cette crise sanitaire, le Gouvernement accorde une augmentation de circonstance aux collectivités, qui ont été complètement oubliées pendant le premier confinement. Quoi de plus normal en définitive ? Elles ont été la seule digue démocratique et efficace qui tenait debout, face à l'État jacobin qui, lui, passait d'En Marche à la déshérence, croulant sous la bureaucratie, l'impréparation et l'incapacité à saisir le réel et à prendre des décisions d'urgence claires, pour finir par sombrer dans la restriction de libertés individuelles, économiques et démocratiques. À long terme, la fiscalité économique locale devient une variable d'ajustement et les collectivités se voient privées durablement de leurs marges de manoeuvre propres. Que les maires en soient ici informés : la diminution de 10 milliards d'euros d'impôts de production est une fausse bonne nouvelle, car ce sont les communes qui vont payer ! Une fois de plus, l'État se montre généreux, mais avec l'argent des autres Pour que cesse la fiscalité confiscatoire, c'est à l'État de prendre ses responsabilités et de réduire son train de vie, car la dépense publique est tournée, non plus vers le citoyen, mais vers l'État lui-même. Pour relocaliser et redevenir compétitif, il faut aussi que l'État accepte une baisse des charges salariales, mais aussi une TVA réduite sur les produits « Made in France ». Ce n'est pas l'Union européenne et son ultralibéralisme qui nous le permettront. C'est cette même Union européenne qui, avec son obsession de l'harmonisation des tarifs, veut que le taux de la taxe sur la consommation finale d'électricité soit centralisé et fixé à son niveau plafond. On a beau dire ce que l'on veut dans cet hémicycle, ce sont les règles de Bruxelles qui s'imposent à chaque échelon de notre organisation territoriale. Incarcérés dans cette geôle européiste que vous appelez Union européenne, vous nous privez de la liberté nécessaire pour insuffler une stratégie incitative d'avenir. Enfin, avec les restrictions que nous vivons encore aujourd'hui dans nos cafés, hôtels, restaurants et dans notre liberté de circuler, ce PLF 2021 devrait prendre en compte les nouvelles dépenses engendrées par la crise sanitaire, devenue crise économique et sociale, dont l'impact atteint les collectivités locales les plus fragiles. On ne donne donc pas assez les moyens aux collectivités de participer à l'effort de relance. Combien faudra-t-il d'échecs et de projets de loi de finances rectificative en 2021 pour que l'on accepte une réforme financière et territoriale en profondeur ? Pour s'administrer librement, encore faut-il que les communes soient libres, et ce n'est pas ce PLF 2021, qui restreint leurs libertés fiscales, qui le leur permettra

madame la ministre, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, depuis le mois de mars, les collectivités locales- qu'il s'agisse des communes, des intercommunalités, des départements ou des régions -sont en première ligne dans cette crise sanitaire sans précédent.

Ce sont elles, aussi, qui ont imaginé des solutions pour prendre en charge les enfants en accueil périscolaire et dans les crèches, ou pour les maintenir à l'école. Ce sont elles, encore, qui ont assuré la tenue des marchés ou appuyé le déploiement des campagnes de tests. Enfin, ce sont leurs services publics de proximité qui demeurent souvent le seul ancrage de la République, en répondant aux besoins quotidiens des habitants. Parallèlement, les collectivités locales subissent une baisse importante de leurs recettes fiscales, domaniales ou tarifaires. L'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité estime ainsi que le coût de la crise sanitaire s'élèvera pour les communes à 8 milliards d'euros sur trois ans, dont près de 6 milliards pour l'année 2020. Quant aux départements, ils vont probablement enregistrer à court terme une forte progression de leurs dépenses sociales, que ce soit pour le financement du revenu de solidarité active (RSA), pour la contribution aux tarifs des Ehpad, ou encore pour le soutien aux associations et aux entreprises. Cette discussion budgétaire s'inscrit donc dans un contexte très particulier, car la crise sanitaire liée au covid-19 frappe douloureusement l'ensemble de nos collectivités territoriales. Aussi, les crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » que nous examinons aujourd'hui doivent être mobilisés plus que jamais au service de nos territoires, d'autant que les inquiétudes des élus locaux sont très importantes. En effet, la baisse des impositions économiques et leur compensation par une part d'impôt national s'inscrivent dans la tendance lourde d'une perte d'autonomie fiscale pour les collectivités territoriales, au travers du remplacement de produits d'impositions sur lesquelles les collectivités disposent d'un pouvoir de taux ou d'assiette par des produits d'impôts nationaux. La suppression de la taxe d'habitation, la baisse de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises (CFE), ou encore, cette année, la réduction de la moitié de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) des finances publiques (DGFiP) de taxes diverses comme celle sur l'électricité donnent aux collectivités territoriales le sentiment de n'être plus que les gestionnaires de dotations de l'État. Nous déplorons donc l'étouffement progressif de leur autonomie financière. Donner aux élus locaux la possibilité d'actionner les leviers fiscaux est un impératif démocratique dans le cadre d'une République pleinement décentralisée.

Concernant plus précisément la mission « Relations avec les collectivités territoriales », c'est avec satisfaction que je constate que ses crédits connaissent une augmentation significative, de l'ordre de 6,82 % en autorisations d'engagement et de 12,88 % en crédits de paiement,

Je souhaite également saluer l'article 57, qui prévoit l'entrée en vigueur progressive de l'automatisation du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). Déjà reportée à deux reprises, cette mesure devrait faciliter sa gestion à tous les niveaux. Nous savons que certaines collectivités étaient remboursées par le

Or le FCTVA constitue l'une des principales aides aux collectivités territoriales en matière d'investissement et un solide levier qu'il convient d'exploiter dans le cadre de la relance économique. J'ai entendu avec plaisir Charles Guené évoquer la redéfinition du FPIC.

Madame la ministre, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, les crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » sont en mesure de contribuer efficacement à la relance et à la transformation de nos territoires. C'est pourquoi le groupe Les

Benarroche. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, nous abordons aujourd'hui l'une des missions qui se tient au coeur de notre assemblée représentante des territoires. d'autorisations d'engagement constituent un levier financier majeur, non seulement dans la péréquation des moyens en local, mais aussi comme levier de l'investissement local, particulièrement en milieu rural, avec les impératifs de la transition écologique. Comme souvent, l'échelon local a su répondre « présent » ces derniers mois en s'adaptant très rapidement aux exigences de la situation. J'en profite pour saluer le milliard d'euros supplémentaire de la dotation de soutien à l'investissement local exceptionnelle attribué par le plan de relance. Mon groupe se félicite d'un fléchage de ces crédits prenant en compte l'empreinte carbone et l'impact sur la biodiversité des projets soutenus. Nous devons transformer l'essai et convertir cela en écoconditionnalité. Il y a un pas supplémentaire que j'encourage le parlons de la biodiversité et des moyens engagés pour la préserver. La dotation « biodiversité », anciennement Natura 2000, est stable et ne représente qu'une faible part du soutien aux projets des communes qui font face à des charges résultant de leur appartenance à une zone protégée, à des parcs nationaux groupe présentera donc un amendement afin de permettre une réévaluation des sommes présentées par le Gouvernement, qui nous paraissent encore éloignées des enjeux. J'ai déjà pu aborder l'importance que nous devrions accorder au maintien d'une gouvernance plus sereine, au développement d'une démocratie plus forte localement cela doit s'accompagner de moyens. La loi relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, qui n'a pas un an, se voit confirmée dans les crédits de ces missions avec la réalisation de quelques avancées : une « protection fonctionnelle », le remboursement des frais de garde et d'assistance des enfants ou des personnes âgées et handicapées pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants. J'espère que les moyens incitant à une plus grande participation des élus locaux pourront se voir étendus à des collectivités de taille plus importante. Nos collectivités restent parfois à la porte de tous ces financements. Je pense notamment à la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR), dont j'entends les objectifs d'une ventilation sur un plus grand nombre de projets. comme le rappelait mon collègue Paulu Santu Parigi, il existe toujours un différentiel important entre les crédits disponibles et les crédits consommés, et les montants disponibles devraient faire l'objet d'une meilleure communication.

Je souhaiterais aborder aussi, dans le cadre du programme 122, « Concours spécifiques et administration », les moyens financiers dédiés aux situations de détresse extrême dans lesquelles peuvent se trouver les communes, principalement ceux qui sont destinés à la réparation des dégâts causés par les calamités publiques. Il n'est malheureusement pas surprenant de constater dans les documents annexes l'augmentation du nombre de dossiers présentant des dégâts de plus d'un million d'euros. Les catastrophes naturelles sont plus nombreuses, et plus dévastatrices. Le changement climatique y est pour beaucoup. Ces 30 millions d'euros sont essentiels pour réparer les dégâts, mais nous restons persuadés qu'une politique budgétaire tournée vers la prévention de ces risques, au travers d'une meilleure prise en compte de la transition écologique dans chaque projet local, est essentielle.

le manque de visibilité des financements et des dotations de l'État peut fortement complexifier le travail de nos communes et des autres collectivités locales. Certes, les lois de programmation financière existent, mais leurs orientations proclamées à échéances irrégulières et changeantes, et l'actualisation permanente de données macroéconomiques ne permettent pas, souvent, de sécuriser les exécutifs locaux dans leur planification budgétaire. Voilà, madame la ministre, monsieur le secrétaire d'État, l'analyse du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires des crédits de cette mission, qui ne semblent pas à la hauteur de la transition écologique, qui doit être entreprise au niveau local, en partie avec le soutien financier de l'État. Porteur de ces attentes des collectivités, notre groupe ne votera pas ces crédits.

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, nous démarrons ce matin l'examen des crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » Cette mission est l'occasion de rappeler le soutien de l'État aux collectivités, mais aussi aux élus locaux, en cette période inédite. Elle s'inscrit dans la continuité des actions que le Gouvernement mène résolument depuis trois ans en faveur des territoires redonner du pouvoir aux élus locaux et les replacer au coeur des territoires ; prévoir une meilleure adaptation des politiques publiques aux spécificités locales ; favoriser la revitalisation des territoires accélérer la transition écologique ; et renforcer la santé financière des collectivités. Sur ce dernier point, au coeur de la crise sanitaire, l'État n'a pas failli et a accompagné les collectivités, notamment par les mesures d'urgence prises lors de la troisième loi de finances rectificative (LFR 3). Nous avons adopté plusieurs mesures d'accompagnement des collectivités lors de la première partie du PLF. Je pense notamment à la garantie des fonds départementaux de répartition des DMTO des petites communes de moins de 5 000 habitants. Concernant la mission RCT, les crédits sont en hausse de 6,9 %, pour un budget s'élevant à 4,1 milliards d'euros pour 2021. Au sein de cette mission, le soutien de l'État aux collectivités se décline en trois axes. Premier axe l'attribution de ressources aux collectivités territoriales pour soutenir les territoires les plus fragiles. La mission prévoit un maintien historique des concours financiers de l'État aux collectivités territoriales pour 2021, avec une dotation globale de fonctionnement (DGF) à 26,8 milliards d'euros pour la quatrième année consécutive, soit 8,3 milliards pour le bloc communal et 8,5 milliards pour les départements. À cela s'ajoutent des variables d'ajustement historiquement faibles de 50 millions d'euros et une accélération du rattrapage de la

pour le remboursement par l'État de l'achat de masques effectué par les collectivités entre avril et juin derniers, et pour l'abondement exceptionnel d'un milliard d'euros supplémentaires pour la DSIL intervenu dans le cadre de la LFR 3. Pour les communes en grandes difficultés financières, des subventions exceptionnelles de fonctionnement peuvent être accordées. Pour l'année 2021, ces subventions s'élèvent à 2 millions d'euros. L'État fait également jouer la solidarité nationale en cas d'événements climatiques ou géologiques de très grande ampleur. Il prévoit l'attribution de subventions pour contribuer à la réparation des dégâts sur les biens des collectivités. En 2021, 40 millions d'euros sont prévus à cet effet. Deuxième axe : l'accompagnement à l'investissement local, notamment en milieu rural, dans une logique de projet. Nos collectivités locales ont besoin que l'investissement local se poursuive. C'est pourquoi cette mission reconduit les montants des dotations d'investissement à un niveau record à plus d'un milliard d'euros, la dotation de soutien à l'investissement local à 570 millions d'euros, la dotation politique de la ville à 150 millions d'euros, la dotation de soutien à l'investissement des départements à 212 millions d'euros. et dernier axe de cette mission : la compensation des charges transférées aux collectivités dans le cadre de la décentralisation ou les pertes de produit fiscal induites par des réformes des impôts locaux. différentes dotations générales de décentralisation (DGD) instaurées par le programme 119 et gérées par la direction générale des collectivités locales. La dotation générale de décentralisation attribuée aux communes et à leurs groupements s'est stabilisée depuis s'élevant en 2021 à 130 millions d'euros. En 2021, les transferts de compétences ont été compensés dans plusieurs domaines, tels que l'élaboration des documents d'urbanisme, le financement des services communaux d'hygiène et de santé, l'entretien de la voirie nationale de la Ville de Paris ou encore les monuments historiques. La dotation générale de décentralisation attribuée aux régions est quant à elle fixée à hauteur de 1 200 milliards d'euros pour 2021. Elle comprend notamment la dotation de continuité territoriale (DCT) attribuée à la Corse, la DGD versée à Île-de-France Mobilités, pour un montant de 128 millions d'euros, ou la régionalisation de l'assiette de TICPE (taxe intérieure de De plus, en 2021, cette action bénéficie de 300 000 euros supplémentaires au profit des conseils régionaux pour la formation professionnelle. Cette mission RCT prévoit également le versement par l'État d'une

La mission RCT traduit le soutien de l'État aux collectivités, mais également aux élus locaux. Afin d'améliorer les conditions d'exercice du mandat des élus locaux, la loi Engagement et proximité prévoit que les membres du conseil municipal bénéficient automatiquement d'un remboursement par la commune des frais de garde d'enfants qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions obligatoires, dans la limite du SMIC horaire. La mission RCT prévoit une enveloppe de 7 millions d'euros à cet effet. Mes chers collègues, nous examinons conjointement à la mission le compte de concours financiers « Avances aux collectivités territoriales » regroupant le produit des impositions locales versé aux collectivités territoriales. Plusieurs éléments sont à noter : 700 millions d'euros sont prévus en 2021 pour les avances de DMTO aux départements ; 111 milliards d'euros d'avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes. Donc, mes chers collègues, la mission RCT et le compte financier « Avances aux collectivités territoriales »

je commencerai mon intervention en saluant le rôle qu'ont joué les collectivités dans la lutte contre la pandémie, que ce soit à travers l'achat de masques à destination de la population ou en termes de soutien aux acteurs économiques. Quand bien même elles n'étaient pas compétentes en matière de santé, les collectivités ont montré que, face à l'urgence, elles pouvaient agir dans les domaines ou l'État est parfois bien moins efficace qu'elles. Si ces actions se sont souvent caractérisées par une hausse de leurs dépenses, leurs recettes se sont également creusées du fait d'une baisse globale de la consommation, mais également d'un report de l'investissement des entreprises. À cela s'ajoute une baisse globale de 10 % des droits de mutation à titre onéreux, mais également le fait que certaines de ces recettes soient perçues avec une ou plusieurs années de décalage ; je pense notamment à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Au total, la perte des collectivités est estimée à près de 6,2 milliards d'euros : de quoi nuancer l'apparente stabilité des finances des collectivités locales, surtout si l'on y ajoute le contexte de perte d'autonomie fiscale par la suppression progressive de la taxe d'habitation depuis 2017. L'idée est non pas de reprendre ce débat, mais d'appuyer sur le fait que la taxe d'habitation était autant un outil qu'un marqueur politique pour de nombreuses collectivités. Sa suppression ne s'est pas faite sans mal pour nombre de communes. Cette mission, si elle est stable, ne retranscrit pas l'ensemble des relations entre l'État et les collectivités territoriales et, en cela, elle porte mal son nom. Si l'on s'en tient aux relations financières, et donc aux concours financiers de l'État, on constate qu'ils atteignent près de 54 milliards d'euros pour 2021, soit une augmentation de presque 4 milliards d'euros. Au sein de ces concours financiers, seulement 8 % des crédits sont alloués à la mission « Relations avec les collectivités territoriales », soit un peu plus de 4 milliards d'euros. Vous le savez, chers collègues, cette mission a deux buts. d'abord, de compenser les transferts de compétences. Cette année, le point notable est la hausse de la dotation générale de décentralisation des régions. Elle vient compenser l'arrêt du versement aux régions des frais de gestion de la taxe d'habitation et respecter le principe d'une dotation égale en 2020. Je m'attarderai plus sur le deuxième but de la mission qu'est le subventionnement aux projets d'investissement dans nos territoires. Si, aujourd'hui, l'essentiel est la lutte contre la crise sanitaire qui nous touche et la réflexion sur un vaccin, il nous faut parer à la crise économique et sociale qui s'abat également sur notre pays. Puisque gouverner, c'est prévoir, nous devons anticiper la relance, qui pour être efficiente devra se faire par les territoires. Le Sénat l'a compris en votant dans la LFR 3 l'ouverture d'un milliard d'euros au titre d'une dotation de soutien à l'investissement local exceptionnelle, tout en permettant que cette enveloppe puisse financer des projets éligibles à la DETR. Cette relance par l'investissement, nous y croyons. Aussi proposerons-nous, par voie d'amendement, de supprimer le seuil de participation minimale de 20 % auquel sont soumises les collectivités maîtres d'ouvrage sur des opérations d'investissement.

À ce titre, nous proposerons, par voie d'amendement, de soutenir davantage les petites communes à dimension touristique, mais aussi d'augmenter la dotation de solidarité rurale de 20 millions d'euros. La crise a prouvé la nécessité d'accès à un service public de proximité ; ce constat doit s'accompagner de moyens importants ; le RDSE y est attaché. Concernant les articles rattachés à la mission, la mise en oeuvre de l'automatisation du fonds de compensation pour la TVA est une mesure de consensus et de simplification des rapports entre l'État et les collectivités ; de ce fait, nous la soutiendrons. Sur l'article 58 et la dotation globale de fonctionnement (DGF), nous constatons, au même rythme que l'année dernière, une légère progression de la péréquation verticale des communes. Nos collègues à l'Assemblée nationale ont esquissé le sujet, mais il nous faudra peut-être à terme réinterroger le fonctionnement de la DGF, qui fait la part belle aux communes urbaines et pénalise les communes rurales et hyper-rurales. Concernant la péréquation horizontale, nous proposerons, par un amendement de notre collègue Christian Bilhac, de répartir le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales à parts égales entre les communes et les intercommunalités, l'objectif étant de renforcer la péréquation en faveur des communes qui en ont le plus besoin.

Demain, les collectivités, communes, départements et régions, auront bien évidemment un rôle à jouer pour sécuriser le bien-vivre de ces femmes et de ces hommes.

je note tout de même que le Gouvernement a fait le choix d'un remboursement partiel des achats de masques effectués du 13 avril au 1 juin. Or nous savons toutes et tous ici que les collectivités locales n'ont pas attendu le 13 avril pour investir dans des masques afin de répondre aux

leur réactivité et de leur agilité pour contribuer au fonctionnement du pays. Qu'aurait été notre pays sans les collectivités, qui ont maintenu des services essentiels et permis la réouverture des écoles ?

seulement 3,6 % du montant des transferts financiers de l'État aux collectivités et 1,6 % du montant global de leurs ressources. En cette période de crise sanitaire, économique et sociale, chacun en convient, les collectivités ont été le premier rempart face aux conséquences de l'épidémie de la covid-19. Elles ont fait preuve de rapidité, achetant des masques dès le début du mois de mars, et d'adaptabilité, répondant aux injonctions parfois contradictoires de l'État, entre confinement et déconfinement, en particulier en matière scolaire. Elles se sont mobilisées pour soutenir les entreprises locales, les commerces et les associations. Elles ont organisé la solidarité, en venant en soutien des personnes âgées et isolées et en distribuant l'aide alimentaire aux plus fragiles. Tout cela s'est traduit par des dépenses supplémentaires imprévues. Dans le même temps, leurs recettes fiscales, domaniales et tarifaires se sont écroulées, à hauteur, selon les estimations, de 5 à 8 milliards d'euros, et ce avant le second confinement. L'effet combiné des dépenses nouvelles et de la chute des recettes a été une dégradation de l'autofinancement, ce qui s'est traduit par un recul de 14 % des dépenses d'investissement. C'est dire que le présent projet de loi de finances était attendu. Malheureusement, il est source, pour les collectivités, de multiples désillusions. Désillusion d'abord sur la faiblesse du dispositif des garanties de ressources introduit au PLFR 3. Après les annonces du Gouvernement assurant de son soutien

Désillusion ensuite sur le refus de compenser les pertes de recettes tarifaires sur les droits de place, la taxe de séjour, les locations de salles ou les recettes de casinos, qui représentent plus de 2 milliards d'euros. également sur la prise en compte insuffisante des dépenses spécifiques à la lutte contre la covid-19, que ce soit sur la date et le montant de prise en charge pour l'achat des masques ou sur l'ensemble des investissements et dépenses de fonctionnement supplémentaires pour maintenir l'accès aux services publics locaux. Désillusion enfin de voir une fois encore la DGF gelée, même si le Gouvernement s'enorgueillit de la maintenir, actant ainsi un nouveau recul- j'y reviendrai. C'est ce moment particulièrement difficile que l'exécutif a choisi pour accélérer le bouleversement de la fiscalité locale. D'abord, il poursuit sa réforme de la taxe d'habitation (TH), en engageant pour un tiers la disparition de la contribution des 20 % des ménages les plus aisés. La réforme nécessitera de trouver 10 milliards d'euros sur les trois années à venir et creusera encore les inégalités au détriment des plus modestes, ceux qui ne payaient pas la TH et qui ne gagnent donc Cette réforme aurait pu être reculée d'une année. Ensuite, il privilégie une politique de l'offre, en diminuant de 20 milliards d'euros sur deux ans les impôts des entreprises, alors qu'une grande partie de nos concitoyens ont vu leur pouvoir d'achat amputé. Dès cette année, les entreprises bénéficient d'une remise de 7 milliards d'euros de CVAE, prélèvement qui, comme son nom l'indique, est une taxe sur la valeur ajoutée, et non un impôt de production, car prélevé en aval du processus de production et adapté à l'activité de l'entreprise. Voilà une offrande à laquelle n'accéderont pas les TPE et PME dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 000 euros. un cadeau qui bénéficiera aux plus grandes entreprises sans aucune contrepartie en termes d'emploi, d'engagement écologique ou d'amélioration des droits sociaux. De même, la taxe foncière et la cotisation foncière des entreprises baisseront de 50 %, pour 3,4 milliards d'euros. La compensation, elle, sera gelée sur les taux de 2020. Mesquinerie supplémentaire, le Gouvernement a décidé de minorer l'évolution des bases des locaux industriels, privant ainsi les collectivités de leur dynamique. Ces décisions, qui étaient discutées au sein du Gouvernement depuis le début du quinquennat, n'ont rien à voir avec la relance. Au contraire : elles pénalisent les capacités d'investissement des collectivités. Elles sont la réactivation d'une vieille lune libérale et de la stratégie du ruissellement. On nous justifie cette réforme par un différentiel de compétitivité avec nos voisins. La France serait « moins attractive », alors que nous sommes le pays qui a accueilli le plus d'investissements étrangers en Europe en 2019. De plus, il faudrait comparer ce qui est comparable et se mettre d'accord sur ce qu'est un impôt de production : ainsi, en Allemagne, le, une variante de la taxe professionnelle, rapporte 50 milliards d'euros aux communes et n'entre pas dans le champ des impôts de production au sens de la comptabilité européenne. Si l'on ajoute à cela la nationalisation des 2,3 milliards d'euros de la taxe locale sur la consommation finale d'électricité, qui ôte au passage aux collectivités la faculté de mener une politique tarifaire en faveur des plus précaires, on assiste à un remplacement de la fiscalité locale par des dotations et à une substitution du contribuable local par le contribuable national. La part de la fiscalité ne représente plus qu'un quart des recettes des collectivités, quand les transferts de l'État sont supérieurs à 45 C'est une très mauvaise nouvelle pour les collectivités, trop averties des conséquences des compensations annoncées à l'euro près qui se traduisent dans la durée par une perte financière. J'en viens aux crédits de la mission et aux articles rattachés. Tout d'abord, si

Madame la ministre, la DGF est devenue illisible, complexe et injuste. Le dispositif a atteint ses limites. Il faut avoir le courage de le réformer. Nous y sommes prêts. L'êtes-vous ? Pour le reste, la DETR est stable. L'Assemblée nationale a apporté des améliorations bienvenues quant à son éligibilité. Mais nous aimerions connaître le niveau d'exécution des crédits de paiement, un certain nombre de communes se plaignant d'attendre fort longtemps le versement des subventions. La DPV ne bénéficie toujours pas d'une réévaluation que nous avions déjà réclamée à la suite de l'élargissement du nombre de communes éligibles en 2017. La DSIL est significativement augmentée en autorisations d'engagement dans la mission « Plan de relance ». Cependant, nous nous étonnons qu'il n'y ait que 100 millions d'euros inscrits en crédits de paiement, alors que de nombreuses opérations pourraient démarrer rapidement. outre, nous réitérons notre souhait que cette dotation soit à la main des préfets de département, dans un souci de simplification, de lisibilité et d'efficacité, notamment par la possibilité de la cumuler avec la DETR. Cela étant, si le bloc communal se satisfait de ces crédits d'investissement, les dotations sont fléchées par l'État sur des priorités définies par lui, alors qu'il serait plus conforme à l'esprit de la décentralisation qu'elles soient libres d'emploi et abondent l'autofinancement. Les départements ont perdu 3,4 milliards d'euros de recettes en 2020 et voient leurs dépenses sociales flamber. Le PLFR 4 prévoit 200 millions d'euros de soutien, mais rien pour 2021, alors que- nous le savons -le RSA va croître de manière exponentielle. Madame la ministre, nous pensons que la question de la recentralisation du financement du RSA doit maintenant être posée. des départements (DSID) reste au même niveau qu'en 2019. Son architecture en deux fractions n'a pas été modifiée, laissant plus des deux tiers de l'enveloppe à la main des préfets sous forme d'appels à projets, alors que, là aussi, elle pourrait utilement abonder l'autofinancement, mis à mal par la crise. crise. Je souhaite lancer une alerte sur le programme concernant les aides aux collectivités victimes de catastrophes naturelles, qui nous semble sous-doté, alors que nous connaissons une multiplication des phénomènes climatiques extrêmes. Autre alerte : si tout le monde se réjouit que soit enfin déclenchée l'automatisation du FCTVA, nous resterons vigilants sur le périmètre de l'assiette,

Après la suppression de la taxe professionnelle, dont on mesure aujourd'hui douloureusement la promesse de compensation à l'euro près, vous accélérez le détricotage de la fiscalité locale, en engageant la suppression totale de la TH et celle de la moitié de la fiscalité des entreprises- et ne doutons pas Vous coupez le lien entre l'impôt, le citoyen, l'entreprise et le territoire. Pourtant, ce lien et le levier fiscal qui en découle sont un impératif démocratique d'une République décentralisée.

l'ensemble de nos collectivités : communes, intercommunalités et départements sont particulièrement touchés par la crise sanitaire que nous traversons. Il était, me semble-t-il, nécessaire, et vous l'avez fait- c'est donc un

c'est avec une attention singulière que nous engageons cette discussion au regard du rôle majeur joué par les collectivités territoriales depuis le début de la crise sanitaire et des besoins immenses qui apparaissent.

les collectivités territoriales pouvaient espérer un budget pour 2021 tirant les leçons de 2020 et une nouvelle ambition, avec des moyens correspondants. Or le PLF pour 2021 entérine au contraire le recul de l'autonomie fiscale des collectivités, plus dépendantes que jamais des choix financiers de l'État.

et pour cause, aussi importantes ! Les déconvenues portent moins sur la dynamique elle-même des crédits- ils sont relativement stables -que sur l'altération des équilibres au sein de la mission, conséquence de la réforme de la fiscalité locale. La disparition de la CVAE pour les régions et la compensation de la taxe d'habitation du bloc communal enlèvent toute dynamique fiscale. Comme l'a relevé notre rapporteur spécial Charles Guené, les régions ne disposeront plus que d'un levier fiscal de 10 alors qu'on leur confie la compétence économique et la relance, les départements de 33 % et les communes d'à peine plus de 60 %. Il y a là un risque réel et historique de rupture du lien entre le contribuable et les collectivités. À cet égard, la suppression par le Sénat de l'article 13 du projet de loi de finances, qui prévoit d'unifier au niveau national les tarifs de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité est à saluer. Une telle mesure aurait entraîné une hausse de la taxation d'électricité pour nos concitoyens et une perte

L'Association des maires de France évalue le cumul des dépenses nouvelles et des pertes de recettes liées à la crise sanitaire à près de 8 milliards d'euros sur trois ans. Autant de moins pour l'autofinancement, donc l'investissement public local ! Ne l'oublions pas, la commune est souvent le premier investisseur sur nos territoires. Le soutien de l'État à l'investissement local la DETR et la DSIL, qui est indispensable à la relance de l'activité économique, n'a de sens que si les collectivités concernées peuvent continuer d'investir et si les conditions de cumul vont au-delà de cas exceptionnels.

! La facture finale ne sera pas neutre pour les collectivités : selon les premières estimations, cette crise leur coûtera 8 milliards d'euros entre 2020 et 2021. Face à cette indéfectible mobilisation des collectivités locales, on aurait pu s'attendre à une forme de reconnaissance budgétaire. Hélas, nos espoirs ont vite été douchés Une fois encore, nous nous retrouvons face à un État ingrat qui demande beaucoup, aide un peu et contrôle excessivement nos collectivités, en bridant leur autonomie. La mise sous tutelle des collectivités se poursuit inexorablement, notamment avec l'étouffement progressif de leur autonomie financière. Après la suppression de la taxe d'habitation, vous revenez encore une fois à la charge cette année. La facture s'allonge pour promouvoir votre politique fiscale : 10 milliards d'euros par an de recettes économiques locales en moins sont à prévoir avec les dégrèvements sur les impôts de production- CVAE et CFE. CFE. Vous faites payer une nouvelle fois aux collectivités locales ces choix unilatéraux qui seront lourds de conséquences. Et permettez-nous de douter de la sincérité d'une compensation « à l'euro près », qui n'a jamais été qu'un supplétif temporaire à la baisse des ressources des collectivités. Non, madame la ministre, monsieur le secrétaire d'État, les budgets des communes ne sont pas des budgets annexes de l'État ! Non, les élus ne sont pas les sous-traitants de la politique nationale ! La libre administration et l'autonomie fiscale des collectivités territoriales sont pourtant deux principes constitutionnels. Les collectivités locales ne sont pas de simples échelons administratifs, et les élus locaux sont des majeurs capables. On n'a jamais autant parlé de décentralisation. Pourtant, les coups de canif portés à l'autonomie des collectivités territoriales ne manquent pas. Le malaise des élus locaux vient de cette situation, où ils se sentent dessaisis de leurs prérogatives, tout en devant répondre en première ligne à des citoyens-consommateurs de plus en plus exigeants et empressés. En outre, comment partager la satisfaction du Gouvernement sur l'état des finances locales et sur l'aide apportée aux collectivités durant la crise ? Les modalités de calcul retenues par le Gouvernement, l'exclusion des recettes tarifaires et l'impossibilité pour certains acteurs, notamment les établissements exploités en régie, d'y avoir droit rendent le dispositif de compensation bien trop limité. Rien sur les pertes tarifaires, alors que des centaines de communes ont vu leurs casinos, leurs campings municipaux et leurs piscines fermer. De même, il y aurait à dire sur les concours de l'État : cette année encore, la DGF reste gelée à son niveau de 2013 et n'intègre ni les effets négatifs de l'inflation ni ceux de l'augmentation de la population. Contrairement à l'État, les communes ne peuvent pas recourir à la dette pour financer leurs dépenses de fonctionnement. Dans ce contexte, leurs capacités d'investissement seront inexorablement écrasées, alors même que les collectivités locales réalisent 70 % de l'investissement Enfin, madame la ministre, monsieur le secrétaire d'État, vous connaissez ma détermination à faire évoluer le mode de calcul du FPIC afin de le rendre moins indigeste pour certaines collectivités, telles que les communes frontalières ou les stations de ski. La période exceptionnelle que nous vivons, marquée par un arrêt brutal de l'activité ski en mars dernier et la fermeture des remontées mécaniques jusqu'au mois de janvier 2021, va engendrer des pertes considérables pour les collectivités montagnardes, bien supérieures aux aides qui leur sont promises. Certaines d'entre elles, confrontées à des charges très lourdes et des enjeux importants, se trouvent aujourd'hui dans une situation très délicate. Au regard de ce contexte, je souhaite que mes amendements et ceux de mes collègues qui visent à mieux prendre en compte la réalité de ces communes dans le mode de calcul du FPIC soient entendus avec plus d'acuité que lors des exercices budgétaires précédents. En cette période de crise aiguë, il convient plus que jamais de soutenir les locomotives de notre pays et, croyez-moi, la montagne en fait partie ! La parole

est à Mme la ministre. Madame la présidente, monsieur le rapporteur général, spéciaux, monsieur le rapporteur pour avis, mesdames, messieurs les sénateurs, Joël Giraud et moi-même sommes heureux d'être avec vous aujourd'hui pour examiner les crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » et les amendements qui y sont rattachés. Comme l'a souligné la présidente de la délégation aux collectivités territoriales, Françoise Gatel,

Comme vous le savez, l'examen de ce budget s'inscrit dans un contexte exceptionnel, dont la première conséquence est de « casser les barrières » entre les différentes lois de finances et les diverses missions.

Vous avez également noté que le débat budgétaire était marqué par la discussion du plan de relance, dans lequel les territoires vont naturellement jouer un rôle majeur. En ce

Ce PLF 2021 confirme d'abord les orientations respectées depuis plus de trois ans, au premier rang desquelles le renforcement des moyens accordés aux collectivités. L'année L'année prochaine, les collectivités recevront même de l'État des moyens plus élevés qu'en 2020, avec une augmentation des concours financiers de 1,2 milliard d'euros, déduction faite des mesures de périmètre.

devrait connaître une progression de 546 millions d'euros l'année prochaine du fait de la très bonne tenue des investissements locaux en 2019 et début 2020.

Votre assemblée a aussi adopté un amendement du Gouvernement visant à garantir les fonds communaux de péréquation des DMTO,

que les collectivités, dont les dépenses sont éligibles au FCTVA l'année de la dépense. À l'heure de la relance, cette simplification me semble bienvenue, notamment pour les petites communes, parfois moins « armées » que les grandes pour les tâches administratives.

cette solidarité étant plus que jamais à l'ordre du jour avec la crise que nous connaissons. Dans le détail, la péréquation augmentera de 220 millions dont 90 millions pour la DSU et la DSR, 30 millions pour la dotation d'intercommunalité et 10 millions pour la péréquation des départements. Cet approfondissement de la solidarité bénéficiera largement aux communes d'outre-mer, dont la trajectoire de rattrapage préconisée par le rapport de Georges Patient et de Jean-René Cazeneuve sera accélérée. accélérée. Un autre axe de ce PLF consiste à adapter, comme chaque année, les mécanismes de répartition des concours financiers pour tenir compte des réformes. En l'occurrence, nous tenons notre engagement de rénover

partie du PLF. Un très grand nombre de mesures financières ont été décidées depuis le début de la crise. Si je fais l'addition toutes les annonces faites depuis mars, l'État a déjà décidé de mobiliser plus de 7,8 milliards d'euros au profit des collectivités locales, sous une forme ou sous une autre- compensation,

et les départements un cadre de travail spécifique sur les finances locales. La première réunion avec le bloc communal se tient ce vendredi.

soit un total de 4 081 026 euros pour 2021 au titre du transfert des routes et autoroutes non concédées de l'État à la métropole, en application de la loi du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité

de 118 787 euros au titre du transfert définitif du domaine public de la Dordogne au syndicat mixte Établissement public interdépartemental de la Dordogne (Épidor)

chargés de la gestion des ports départementaux et des ports d'intérêt national, en application de la loi du 13 août 2004.

M. Didier Marie. La crise sanitaire et sociale que nous connaissons a frappé durement bon nombre de nos concitoyens, en particulier ceux qui connaissaient déjà des difficultés. Un million de Françaises et de Français sont ainsi passés sous le seuil de pauvreté. La plupart de ces personnes habitent dans les quartiers prioritaires de la

Les contraintes liées au fonctionnement de cette dotation alourdissent la gestion de ces crédits. La répartition par enveloppe départementale tend à creuser les inégalités entre territoires selon les préfectures chargées de les répartir. le nombre de communes éligibles à la DPV a été élargi, sans que le montant de la dotation soit augmenté. Cela a pour effet de mettre en difficulté les communes les plus précaires. Les communes de métropole et d'outre-mer présentant des dysfonctionnements urbains doivent également faire face à la gestion de la crise sanitaire.

les crédits de la dotation politique de la ville afin de tirer les conséquences de l'élargissement de ses critères d'éligibilité en loi de finances pour 2019. en vertu de l'article 259 de cette loi, le fait de figurer parmi les premiers d'un classement établi en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges composé du potentiel financier par habitant, du revenu par habitant et de la proportion de bénéficiaires d'aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ne constitue plus une condition d'éligibilité à la DPV.

PLF s'élèvent à 90 millions d'euros ; je m'en réjouis. Cependant, ces crédits ne permettent pas un rattrapage de la DSR. L'objet de cet amendement est de contribuer à rééquilibrer la péréquation communale entre les territoires défavorisés, qu'ils soient urbains ou ruraux, sans diminuer les ressources de la DSU.

pour l'année 2021. La dotation biodiversité, anciennement dénommée Natura 2000, permet de soutenir des territoires constitués de sites naturels, terrestres et marins, pour assurer la survie à long terme des espèces et des habitats menacés.

le Gouvernement n'a pas prévu d'augmenter les crédits pour 2021, alors que la préservation de notre biodiversité et des espèces protégées doit être au centre de nos priorités. Parallèlement, le périmètre de la dotation a été étendu aux communes situées au coeur d'un parc naturel ou d'un parc naturel marin.

sont affectés sur les plages du littoral français pour secourir les personnes en danger, réprimer les infractions, traiter les délits de droit commun, ainsi que conseiller les élus locaux. Dans son rapport de 2012, la Cour des comptes soulignait le rôle majeur de ces agents, compétents pour prévenir les noyades des vacanciers comme pour lutter contre la délinquance du sable. sable. Ils n'ont jamais cessé de s'adapter à l'actualité, en luttant dès 2016 contre la menace terroriste, omniprésente sur notre territoire, ou en faisant respecter cette année les recommandations gouvernementales pour lutter contre la pandémie. Malheureusement, en dépit de ce constat, le déploiement des MNS-CRS reste incertain. Si, en 2002, ils étaient 720 à être recensés par la direction générale de la police nationale, pour une présence moyenne de trois mois sur les plages françaises, ils ne sont plus en 2020 que 295 déployés dans soixante communes, pour deux mois de saison estivale. Dans un contexte sécuritaire plus sensible, ce modèle devrait être généralisé à l'ensemble des communes dotées de plage, alors qu'il existe aujourd'hui de grandes disparités d'intervenants.

étant donné que les communes ont à leur charge de rembourser les frais de mission et de déplacement occasionnés par la participation des maîtres-nageurs sauveteurs à la sécurisation des plages des littoraux français. Je me tourne donc cette année vers vous, madame la ministre, monsieur le secrétaire

au FCTVA. Ce fonds obéit à des règles très précises. En l'occurrence, certaines dépenses d'entretien de voirie et de bâtiments publics

lorsque vous faites des travaux d'enfouissement de lignes téléphoniques, qui, souvent, sont dans la même veine et interviennent à la même période, vous ne récupérez pas la TVA et vous êtes obligés de la mettre en frais de fonctionnement. Il y a donc une anomalie dans le système. Au-delà, je trouve qu'il y a beaucoup de flou, d'imprécisions, contrairement à ce que disait mon ami et collègue Charles Guené, dans le système de remboursement de la

Le fiscaliste que je suis estime que l'on doit suivre au maximum les règles qui sont propres à la TVA. Effectivement, dans ce domaine, il y a un flou.

le sais bien, le cas échéant, les dépenses afférentes sont inscrites en section de fonctionnement. Elles ne peuvent donc pas, bénéficier du FCTVA. En revanche, je pense qu'il y a quand même,

L'interprétation des services fiscaux que vous mentionnez dans l'objet de votre amendement, c'est en fait le cas où la collectivité agit en tant que prestataire de l'opérateur, ce qui veut dire qu'elle refacture la totalité des travaux

Le retour de TVA doit se faire au bénéfice des collectivités, car il n'existe pas de refacturation à 100 % de ces travaux à un opérateur. Au mieux, les opérateurs apportent une petite contribution, mais on est loin des 100 %.

en nuage- ou, pour ceux qui parlent le breton. Les échanges entre les rapporteurs spéciaux et l'administration ont permis d'établir que ces dépenses seraient bien intégrées dans l'assiette

Quel est l'avis du Gouvernement ? Les dépenses du seront éligibles de manière automatisée au FCTVA, grâce à la création d'un compte spécifique, dont les caractéristiques seront précisées dans un arrêté qui doit paraître d'ici au 1 janvier.

Il est, de mon point de vue, relativement injuste, voire peu moral que l'État perçoive des recettes de TVA sur ce type de dépenses, c'est-à-dire, d'une certaine manière, sur la misère, et que le contribuable local contribue au financement du budget de l'État. Vous allez me dire que le contribuable local, c'est aussi le contribuable national :

de cet amendement voudraient rendre éligibles au FCTVA les dépenses d'achat d'équipements de protection contre la covid-19. Ce sujet a déjà été examiné en LFR, et l'amendement a été rejeté. Les dépenses

qui n'enrichissent pas le patrimoine de la collectivité. Par ailleurs, et c'est cela qui est important, l'État a déjà mis en place un fonds permettant d'accompagner l'achat des masques par les collectivités, en finançant la moitié de leur coût, après déduction des éventuels autres financements, afin de préparer la sortie du confinement de mai dernier. L'État va ainsi rembourser 215 millions d'euros. J'y insiste, puisque, quand cela avait été décidé, on avait évalué le coût à 60 millions

le rapporteur spécial de la commission des finances, il ne me semble pas que ce soit un bon vecteur pour faire cette opération.